Monsieur le président, madame la ministre,mes chers collègues,le présent projet de loi de finances pour 2018 constitue une traduction du plan Climat, même s'il manque de cohérence sur certains aspects et paraît en deçà des ambitions politiques affichées par le Gouvernement. S'agissant des moyens budgétaires, je relève plusieurs

Madame la ministre, je n'adhère pas à cette nouvelle version de la vision punitive de la fiscalité énergétique portée votre gouvernement qui se traduit par l'accélération de la trajectoire carbone et la convergence par le haut des fiscalités de l'essence et du gazole. D'abord, je regrette profondément que les évolutions du financement des opérateurs proposées dans le projet de budget aient pour trait commun de constituer

de son financement. Or l'augmentation de son budget sera presque totalement absorbée par le règlement des restes à payer issus des engagements passés ! J'ai eu l'occasion de dire que vous n'en étiez pas responsable ; vous en êtes cependant Comment pouvez-vous, dans ce contexte, affirmer soutenir le développement de la chaleur renouvelable et de la politique de prévention et de valorisation des déchets ? De même, la suppression des subventions aux opérateurs de la biodiversité permet à l'État de faire des économies sur le dos des agences de l'eau, qui financeraient, dès 2018, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et l'Agence française pour la biodiversité. Votre gouvernement, madame la ministre, propose de doubler la contribution des agences de l'eau en 2018, ce qui va totalement à l'encontre du principe de la redevance, selon lequel l'eau paye l'eau. L'Agence française pour la biodiversité n'est même pas gagnante, puisqu'elle va devoir reverser une partie de la contribution acquittée par les agences de l'eau aux parcs nationaux. Circuit court, ou court-circuit ? Vous nous donnerez certainement la réponse ... Comme si cela n'était pas suffisant, votre gouvernement prévoyait initialement de diminuer le plafond des recettes affectées aux agences de l'eau.

près de 8 milliards d'euros en 2018, soit une hausse de 10 % par rapport à 2017, principalement due à l'augmentation du coût du soutien aux énergies renouvelables électriques en raison du très fort dynamisme de la filière photovoltaïque. Les projections réalisées par la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, montrent que ces charges s'élèveront à plus de 10 milliards d'euros en 2022, soit 2,2 milliards de plus qu'en 2018, et que le total cumulé atteindra 44,9 milliards d'euros sur la période 2018-2022.

« Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale », dit aussi FACE, le montant des aides versées aux autorités organisatrices de la distribution d'électricité pour le financement des travaux d'électrification en zone rurale diminuera de 4,5

uniformément et aveuglément, les choix. Ce non-choix aura des conséquences pour les territoires ruraux, puisqu'ils seront moins en mesure d'accompagner leur développement démographique et économique en matière de réseaux électriques.

sur le vote des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », et lui propose d'adopter les crédits des comptes d'affectation spéciale « Transition énergétique », « Aides à l'acquisition de véhicules propres »

la ministre. Ce constat a conduit le Président de la République à annoncer une « pause » en matière d'infrastructures de transport, ce qui s'est notamment traduit par une révision à la baisse de quelque 800 millions d'euros des dépenses initialement prévues pour l'AFITF en 2018, les engagements concernés ayant été repoussés à une date ultérieure.

L'équilibre financier de l'AFITF demeurera néanmoins précaire avec des restes à payer en augmentation, s'établissant à 12,3 milliards d'euros,

La taxation des poids lourds étrangers en transit, qui endommagent notre réseau routier sans participer à son financement, demeure une piste que nous devons creuser. Pourrez-vous nous donner, madame la ministre, des informations complémentaires sur l'avancement de ce dossier, dont vous avez annoncé qu'il serait étudié conjointement par le Gouvernement, les régions et le Parlement

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vais vous présenter le programme 159, « Expertise, information géographique et météorologie », ainsi que le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens Concernant Météo France, la subvention pour charges de service public portée par le programme 159 connaîtra, pour la sixième année de suite, une diminution en 2018, pour s'établir à 188,8 millions d'euros. Dans le même temps, ses effectifs diminueront de 95 équivalents équivalents temps plein travaillé, ou ETPT, mouvement qui devrait se poursuivre dans les cinq ans à venir. Si ces suppressions de postes obéissent à une véritable logique et et visent à tirer parti des multiples applications du numérique dans le domaine de la météorologie et de la réorganisation du réseau territorial de Météo France qui s'est achevée à la fin de l'année 2016, il convient toutefois de rester très vigilant pour ne pas affaiblir un opérateur qui joue un rôle essentiel pour la sécurité des personnes des personnes et des biens face à la multiplication des événements climatiques extrêmes. Pour rester un opérateur météorologique de rang mondial, Météo France devra rapidement se procurer un nouveau supercalculateur susceptible de multiplier par cinq sa capacité de calcul. Si les bénéfices socio-économiques de cet outil sont estimés au minimum à douze fois la valeur de cet investissement, l'établissement n'a pas encore obtenu de l'État les crédits nécessaires à son financement, crédits évalués à 100 millions d'euros, dont 55 millions d'euros dans les cinq ans à venir. C'est un sujet qu'il faudrait rapidement L'Institut national de l'information géographique et forestière, l'IGN, verra lui aussi sa subvention pour charges de service public diminuer en 2018, à 91,7 millions d'euros, et ses effectifs perdre 35 ETPT. Mais alors Mais alors que Météo France semble en mesure de voir ses recettes commerciales rebondir à compter de 2017, celles de l'IGN sont sévèrement fragilisées par l'avènement de l'open data et pourraient se réduire comme peau de chagrin dans les années à venir. Il est indispensable que soit menée une véritable réflexion,

alors même que ce regroupement de onze entités préexistantes est âgé d'à peine trois ans dans sa forme actuelle. Le Gouvernement prévoit de lui appliquer tout au long de la législature des réductions de subvention pour charges de service public- atteindra 206 millions d'euros en 2018 -et d'effectifs- 103 ETPT en moins en 2018 -, sans lui offrir pour le moment la moindre perspective, ce qui a conduit, du reste, le président de son conseil d'administration à démissionner. S'il est clair que l'avenir de cet opérateur passe par une collaboration beaucoup plus intense avec les collectivités territoriales, le Gouvernement devra rapidement exprimer ce qu'il attend de lui et cesser de le percevoir uniquement comme une variable d'ajustement, ce qui a été le cas durant de longues années. J'en viens à présent au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », dit BACEA, qui porte les 2,2 milliards d'euros de crédits de la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC. Il est exclusivement financé par le secteur du transport aérien. Dès lors, l'évolution du trafic et la bonne santé des compagnies françaises ont une influence décisive sur son équilibre financier. Le trafic aérien bénéficiera d'une croissance comprise entre 5,4 % et 5,9 % en 2017-

depuis deux ans et si le lancement de la nouvelle compagnie Joon paraît constituer un beau succès pour sa nouvelle direction, qui a su démêler l'écheveau des relations sociales et réarmer industriellement le projet de la compagnie, la compétitivité des compagnies aériennes françaises devra faire l'objet d'un examen attentif. Je salue, à cet égard, l'initiative de Mme la ministre de réunir des assises du transport aérien au premier semestre 2018. Je souhaite que nous puissions progresser à cette occasion sur les thèmes de la compétitivité du transport aérien français. Dans cette conjoncture très favorable, la DGAC bénéficiera de recettes quasiment identiques à celles de 2017, soit un montant légèrement supérieur à 2 milliards d'euros. Cette relative stabilité s'explique notamment par la baisse de 26 millions d'euros des recettes de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole, la RSTCA-M, accordée aux compagnies au départ et à l'arrivée des plateformes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, en contrepartie de l'affectation au BACEA de l'intégralité des recettes de la taxe de l'aviation civile. Je suis heureux de voir que cette mesure favorable au secteur aérien français, que j'avais défendue au Sénat, est à présent entrée en vigueur : il a fallu suivre le dossier de près celles de la redevance de route, les recettes de la taxe de l'aviation civile seront dynamiques en 2018. L'exonération à 100 % de cette taxe pour les passagers en correspondance, que nous avions là aussi adoptée pour aider les compagnies aériennes, a représenté 77,4 millions d'euros d'économies en 2016 pour les compagnies assujetties à la taxe, dont 57 millions d'euros pour Air France. Comme en 2017, le schéma d'emplois pour 2018 de la DGAC ne prévoit pas de suppression d'emplois. Sa masse salariale augmentera de 1,3 % pour atteindre 923,5 millions d'euros. Sur cette somme, 17,7 millions d'euros correspondent aux mesures catégorielles prévues pour 2018 par le protocole social 2016-2019 de la DGAC, dont le coût global représente 55 millions d'euros sur la période, contre 27,4 millions d'euros pour le protocole social 2013-2015 La DGAC maintiendra en 2018 son effort d'investissement porté à 250 millions d'euros par an, auxquels s'ajoutent 50 millions d'euros de fonds de concours européens, de concours européens, depuis 2014. Sur cette somme, 135 millions d'euros sont consacrés à de grands programmes de modernisation du contrôle de la navigation aérienne, dont le coût total représente quelque 1 660 millions d'euros et auxquels je consacre actuellement un contrôle budgétaire. Après une année 2017 difficile, le nouveau gouvernement a décidé de rebudgétiser les crédits consacrés par les deux premiers programmes d'investissement d'avenir à la recherche et développement en matière aéronautique civile pour un montant de 135 millions d'euros de crédits de paiement, ce qui me satisfait.

Monsieur le président,madame la ministre,mes chers collègues,en matière d'énergie, les sujets d'inquiétude ne manquent pas. C'est d'abord l'explosion de la fiscalité énergétique, une tendance de fond des dernières années que ce projet de budget accentue encore, en accélérant la trajectoire de la taxe carbone et en faisant converger, uniquement à la hausse, les tarifs del'essence et du gazole. La commission des affaires économiques est bien entendu favorable à une tarification forte du CO2 qui oriente les investissements vers les énergies bas carbone. Mais nous exigeons, dans le même temps, que cette fiscalité soit non pas punitive, mais véritablement incitative : en clair, que ces hausses soient compensées, comme le prévoit la loi, par une baisse équivalente d'autres taxes. Or nous en sommes très loin Face aux 3,7 milliards d'euros de recettes supplémentaires qu'encaissera l'État, les contreparties annoncées, la prime de conversion des véhicules et le chèque énergie, ne permettront au mieux de restituer Sur les deux prochaines années, la pression fiscale, qui pèsera tout particulièrement sur les ménages modestes et ruraux, augmentera de 3,5 milliards d'euros en 2018, et de 6,1 milliards en 2019 Sous couvert de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, le Gouvernement ne poursuit, en réalité, qu'un unique objectif de rendement budgétaire. Deuxième sujet de préoccupation : le devenir des territoires à énergie positive, dont le financement n'est aujourd'hui pas assuré au-delà de 2018. Compte tenu des 75 millions d'euros supplémentaires annoncés en loi de finances rectificative, l'impasse financière pourrait encore atteindre un maximum de 275 millions d'euros. Même si la responsabilité du trou incombe au précédent gouvernement, il est essentiel que la parole de l'État soit tenue Troisième sujet d'inquiétude : la réforme du crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, reste trop brutale malgré les aménagements prévus par l'Assemblée nationale. des affaires économiques a jugé qu'il serait préférable, pour les chaudières au fioul à haute performance, ainsi que pour les fenêtres en cas de remplacement d'un simple vitrage, de pérenniser un taux réduit à 15 %. Les fenêtres sont en effet un point d'entrée dans un parcours de rénovation, tandis que l'exclusion des chaudières au fioul mettrait fin au renouvellement d'un parc vieillissant et émetteur de gaz à effet de serre, à l'opposé de l'objectif poursuivi.

Plus globalement, la façon dont nous devons examiner les dépenses de soutien aux énergies renouvelables reste très insatisfaisante. Alors que les contrats engagent la collectivité sur des dizaines d'années, le Parlement n'en ratifie que la « tranche annuelle », sans pouvoir débattre des engagements de long terme, et encore moins exercer un véritable contrôle. Les sommes en jeu sont pourtant considérables puisque les appels d'offres lancés depuis 2011 représenteront 65 milliards d'euros de soutien public sur la période 2018-2046. Il est donc urgent de revoir nos procédures d'autorisation budgétaire et d'aller vers la discussion d'une loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, pour redonner toute sa place au Parlement. Tous ces sujets ont conduit la commission des affaires économiques à donner un avis défavorable sur les crédits. La parole

l'adoption des crédits consacrés aux transports routiers figurant dans le projet de loi de finances pour 2018 et dans le budget prévisionnel de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, l'AFITF. Avec les assises de la mobilité qui sont en cours, le Gouvernement veut définir une nouvelle stratégie pour les transports, qui mettra l'accent sur les transports du quotidien et la régénération des réseaux existants. Ces travaux doivent aboutir à la présentation d'une loi de programmation des infrastructures au début de l'année 2018. Nous souhaitons que cette loi tende avant tout à rétablir la soutenabilité du financement des infrastructures et qu'elle permette d'associer davantage le Parlement à la définition de ces dépenses, alors que notre noble assemblée a, en général, peu de visibilité sur le volet « dépenses » du budget de l'AFITF, qui n'est adopté qu'en décembre. J'appelle d'ailleurs de mes voeux la désignation rapide du président de cette agence, pour remplacer Philippe Duron, qui a dû la quitter en juin dernier. Le budget d'intervention de l'AFITF, qui passera de 2,2 à 2,4 milliards d'euros en 2018, reste encore contraint. Il ne peut en effet être considéré comme suffisant que si l'on accepte le fait que l'agence retarde certains paiements, comme elle l'a fait par le passé. Mais dans ce contexte budgétaire tendu, nous pouvons tout de même saluer l'augmentation annoncée de 100 millions d'euros des crédits d'entretien et de modernisation du réseau routier national non concédé. Ces crédits atteindront au total 800 millions d'euros, en comptant les crédits de l'AFITF et ceux de l'État. C'est une vraie nécessité, mais il n'est pas certain que cette augmentation soit suffisante pour enrayer la dégradation du réseau observée depuis quelques années en raison d'une baisse des crédits, mais aussi de l'allongement des délais de rénovation des voiries.

Cette prime a en effet l'avantage d'agir directement sur le parc roulant ancien. Par ailleurs, le recentrage du bonus sur les véhicules électriques a l'avantage de favoriser une filière d'avenir, en pleine émergence. en pleine émergence. Pour l'ensemble de ces raisons, et dans l'attente de la loi d'orientation sur les mobilités annoncée pour le début de l'année 2018 qui doit permettre de résoudre un certain nombre de difficultés,

a constaté que le budget proposé pour les transports ferroviaires, collectifs et fluviaux est un budget de transition- une expression souvent employée par Mme la ministre -, dans l'attente de la réorientation de la politique des transports souhaitée par le Gouvernement. Cette démarche, engagée dans le cadre des assises de la mobilité et du Conseil d'orientation des infrastructures, est positive, car nous ne pouvons plus continuer, comme par le passé, à promettre la réalisation de projets d'infrastructures sans nous assurer de leur faisabilité financière. Il faut donc redéfinir les priorités et en garantir le financement. Ce sera l'objet de la loi de programmation que le Gouvernement a annoncée. se félicite également de l'accent mis sur les transports du quotidien ainsi que sur l'entretien et la modernisation des réseaux existants, dont l'état est très préoccupant, en particulier dans le domaine ferroviaire. En attendant ces évolutions, le budget prévu pour 2018 devrait conduire l'AFITF à retarder certains paiements, comme les années précédentes. Malgré ce contexte budgétaire contraint, vous nous avez rassurés, madame la ministre, sur le respect des engagements de l'État concernant le financement des matériels roulants des trains d'équilibre du territoire, dans les deux régions où il était décalé, le Centre-Val de Loire et les Hauts-de-France. Je souhaiterais Je souhaiterais néanmoins évoquer un dernier sujet d'inquiétude : la situation de Fret SNCF. La Cour des comptes vous a alertée sur ce sujet en juillet dernier, madame la ministre, dans un référé sur le fret ferroviaire. Fret SNCF est pénalisé par le coût et le régime de travail de ses agents, et accumule les pertes. Son endettement croît dangereusement : il faut donc réagir, et vite. Quelle réponse comptez-vous y apporter Pour conclure, afin de rester dans le temps qui m'a été imparti, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui suivra avec attention les travaux relatifs à la loi d'orientation sur les mobilités et à la libéralisation du transport ferroviaire de voyageurs, a émis un avis favorable sur l'adoption des crédits consacrés aux transports ferroviaires, collectifs et fluviaux.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à excuser notre collègue Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui ne pouvait malheureusement être présente aujourd'hui. Nous examinons les crédits relatifs aux transports aériens dans un contexte favorable : le secteur aérien est porté par une croissance robuste sur le plan mondial comme national, dont profitent les compagnies aériennes, les exploitants d'aéroports et l'industrie aéronautique. Après les turbulences traversées en 2016, du fait d'un contexte sécuritaire marqué par les attentats terroristes, la croissance du trafic aérien national a repris avec vigueur en 2017, puisqu'elle a atteint 5,9 % au cours du premier semestre de cette année. Cette croissance du trafic, couplée à un prix du pétrole qui reste faible, permet aux compagnies aériennes françaises de voir leur situation économique et financière s'améliorer. Sur les neuf premiers mois de l'année 2017, le résultat d'exploitation d'Air France a ainsi progressé de 220 millions d'euros. Le lancement, cet été, de la nouvelle compagnie Joon par Air France témoigne aussi de ce dynamisme retrouvé, dont nous pouvons nous féliciter. Cependant, ces évolutions positives ne masquent pas la fragilité persistante des compagnies aériennes, qui continuent de souffrir d'un différentiel de compétitivité vis-à-vis de leurs concurrents, et tout particulièrement des compagnies du Golfe et des compagnies à bas coûts. Ces problèmes de compétitivité, nous en connaissons la cause il s'agit des écarts de charges salariales, du poids de la fiscalité applicable au secteur aérien, ainsi que de la complexité des normes administratives. En cas de retournement de la conjoncture, notamment de remontée rapide des prix du pétrole, ces écarts de coûts pourraient fortement pénaliser le pavillon français. Les prochaines assises du transport aérien devront par conséquent être l'occasion de prendre de nouvelles mesures de soutien à la compétitivité de ce secteur. Un autre sujet d'interrogation concerne la possible privatisation d'Aéroports de Paris, qui soulève des difficultés juridiques, financières et stratégiques non négligeables, et qui pourrait fragiliser le groupe aéroportuaire, alors même que ce dernier est engagé dans d'importants projets de modernisation et de développement du parisien. S'agissant, pour finir, du budget annexe « Contrôle et exploitations aériens », la commission se félicite de la poursuite, en 2018, du désendettement de la DGAC, la direction générale de l'aviation civile, qui conduira à ramener le niveau de la dette à un niveau inférieur à celui d'avant la crise de 2009. La hausse des recettes d'exploitation, du fait de la croissance du trafic aérien, permettra à la DGAC d'assainir sa situation financière, tout en maintenant ses efforts d'investissement pour moderniser les systèmes de gestion de la navigation aérienne. C'est pour cette raison que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis favorable sur l'adoption des crédits relatifs aux transports aériens. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, Charles Revet, rapporteur pour avis, m'a demandé de le remplacer pour émettre l'avis de notre commission. Madame la ministre, notre avis est défavorable tant notre inquiétude est grande sur l'inadéquation des moyens proposés quand on constate le manque de performance des grands ports français, alors que nous avons le deuxième territoire maritime du monde. Trop de structures se superposent- structures d'État, structures régionales, structures de façade, comités de toutes sortes -, ce qui n'est pas de nature à fluidifier les choses ni à faciliter les projets. La gouvernance des ports repose souvent sur une approche trop technique et pas assez économique. Les ports sont dans une situation délicate. Ils perdent des parts de marché par rapport aux autres ports européens. Intégrer une desserte efficace de leur est un élément essentiel de compétitivité. Mais les infrastructures ferroviaires et fluviales ne permettent pas d'acheminer d'une façon performante les marchandises vers les ports de manière fiable, rapide et régulière. L'écluse de Méricourt dans les Yvelines menace de tomber en panne, ce qui bloquerait tout trafic sur la Seine. Exact ! Ce trafic serait transféré sur la route, et il serait bien difficile que le transport fluvial le récupère. Car là aussi il y a besoin de stabilité et de confiance de la part des opérateurs. Pour sauvegarder ces ouvrages, ce sont 100 millions d'euros par an sur dix ans qu'il faudrait prévoir. De même, le développement de l'intermodalité nécessite de gérer le surcoût engendré par les manoeuvres de manutention pour le ferroviaire et le fluvial. Le port de Dunkerque a mutualisé ses coûts ; le résultat semble intéressant.

Vous l'avez rétablie avec l'appui du Premier ministre, par la suppression de l'article 53. Mais enfin, de quel droit une administration, fût-elle de Bercy, se permet-elle en catimini de revenir sur une décision très majoritaire du Parlement ? du Parlement ? L'intervention de M. le Premier ministre au Havre, il y a quelques jours, dans le cadre des assises de l'économie de la mer, a donné espoir à tous ceux qui attendent une véritable politique de développement de l'économie de la mer. Nous serons vigilants à ce que les espoirs ne soient pas déçus. Mais pour le moment et dans l'attente, nous nous prononcerons sur ce qui est factuel, le budget pour 2018. Le budget présenté aujourd'hui dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018 ne permet pas de répondre au risque de décrochage pérenne des ports français ni de mettre en place une politique maritime ambitieuse. Notre commission a donc émis un avis défavorable sur l'adoption des crédits du projet de loi de finances pour 2018 consacrés aux transports maritimes.

Monsieur le président,madame la ministre, mes chers collègues, dans un contexte de changement climatique, de vieillissement des installations industrielles et de mutations technologiques rapides, la politique de prévention des risques revêt une importance croissante. Les moyens qui lui sont dédiés sont donc indispensables, sans qu'il soit possible de transiger avec des missions d'une telle importance pour la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. durable a relevé que les crédits dédiés à la prévention des risques technologiques, miniers, naturels et sanitaires seront globalement préservés en 2018. Toutefois, ce budget témoigne davantage d'un effort de priorisation des actions à moyens contraints que d'un véritable souffle nouveau en faveur de la prévention des risques. L'augmentation des ressources consacrées à la recherche en matière de santé-environnement nous semble opportune, car il s'agit bien d'améliorer la connaissance et la maîtrise des risques sanitaires d'origine environnementale, comme les perturbateurs endocriniens. Dans ce même domaine, le renforcement annoncé des moyens de l'ANSES, en faveur de l'évaluation des produits phytosanitaires nous semble essentiel, compte tenu de l'importance prise par ces sujets dans le débat public, comme l'actualité des derniers jours nous l'a encore rappelé. Quant à l'ADEME, le montant élevé des crédits de paiement permettra d'abord, comme l'a rappelé notre collègue Jean-François Husson, de couvrir d'importants restes à payer accumulés les années précédentes, tandis que la capacité d'engagement de l'agence va diminuer à partir de 2018. À ce titre, la commission a regretté l'absence de revalorisation du Fonds chaleur, dont les ressources sont notoirement insuffisantes pour atteindre les objectifs de la transition énergétique. Deux points de vigilance ont été relevés par la commission. Premièrement, les ressources attribuées à la sûreté nucléaire demeurent sous tension. Or il s'agit d'une mission hautement prioritaire, presque régalienne, de l'État, compte tenu du prolongement du parc existant et de la multiplication des tâches. Il faut également évoquer la découverte, en 2016, d'irrégularités dans la fabrication de certaines pièces de réacteur. Face à la multiplication des enjeux à venir, il faut établir une trajectoire de financement crédible et pérenne pour la sûreté nucléaire de notre pays. Je l'ai déjà dit l'année dernière, il faut repenser totalement le système de financement de la sécurité nucléaire. Deuxièmement, le changement climatique va multiplier les risques naturels de grande ampleur. À cet égard, plusieurs membres de la commission se sont inquiétés du plafonnement des ressources affectées au fonds Barnier par le projet de loi de finances. Le Sénat a adopté en première partie un amendement visant à revenir sur cette décision. Le niveau d'intervention de ce fonds devrait être réévalué pour soutenir les collectivités dans leurs études et travaux, en particulier pour la prévention des inondations. Avec l'indulgence que l'on peut accorder à un premier budget et sous ces différentes réserves, la commission de l'aménagement du territoire

avis. Monsieur le président,madame la ministre, mes chers collègues, j'ai l'honneur d'être rapporteur pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable des crédits des politiques de biodiversité, d'expertise en matière de transition écologique et enfin de transition énergétique.

Le premier point concerne les agences de l'eau. Nous avons déjà eu l'occasion d'en débattre lundi lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, et je me félicite d'ailleurs de l'adoption de l'amendement du rapporteur spécial de la commission des finances qui a supprimé

augmentée cette année à 200 millions d'euros, mettait en péril le budget des agences pour 2018. À trop leur demander d'efforts, les agences ne pourront pas accomplir l'intégralité de leurs missions ô combien importantes, et ce sont les collectivités territoriales qui en seront les premières victimes. Néanmoins, sur la question essentielle de l'eau, je salue l'initiative d'organiser des assises de l'eau en 2018, et je souhaite vivement que le Sénat y soit pleinement associé. Le deuxième point d'inquiétude porte sur la création des premières agences régionales de la biodiversité au début de 2018. Nous devrons prendre garde à ne pas créer de système à deux vitesses en la matière, avec des territoires beaucoup plus avancés que d'autres pour la mise en oeuvre de cette politique de protection de la biodiversité sur nos territoires de métropole et d'outre-mer. Le troisième point concerne le financement des projets des collectivités lauréates de l'appel à projets « territoires à énergie positive pour la croissance verte La circulaire du ministre pointe une « impasse de financement de 350 millions d'euros » ; le précédent Gouvernement rétorque que des crédits auraient dû être prévus cette année ; et le Gouvernement actuel tente de s'en sortir en débloquant 75 millions d'euros dans le projet de loi de finances rectificative.

par avance, madame la ministre, pour vos précisions et les engagements que vous pourrez prendre sur ces sujets importants. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, si j'interviens en tant que membre du groupe Union Centriste sur le temps imparti à mon groupe, je le fais avant tout en tant que président

Nous venons d'entendre pas moins de six rapporteurs qui se sont exprimés sur cette mission. Quatre rapporteurs ont exprimé un avis favorable aux crédits examinés, un rapporteur un avis défavorable, et un a suggéré l'abstention. Cela témoigne de l'approche pragmatique du Sénat et d'un jugement plutôt positif de notre assemblée sur les crédits proposés. Les rapporteurs nous ont éclairés avec beaucoup de précision sur les priorités du Gouvernement en matière d'environnement et de mobilité.

Première observation : ce budget s'inscrit dans le cadre du plan en faveur du climat adopté par le Gouvernement au mois de juillet dernier, lui-même destiné à permettre le respect des engagements pris par notre pays dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Ce plan est ambitieux puisqu'il vise la neutralité carbone en 2050, la fin de la vente de voitures émettant des gaz à effet de serre, la disparition des passoires thermiques, le développement de l'économie circulaire et l'essor des énergies renouvelables. Si nous partageons ces objectifs, leur concrétisation n'apparaît pas encore parfaitement dans ce budget. Certes, nous nous réjouissons que les crédits de la mission soient globalement en hausse, puisqu'ils augmentent d'un peu plus de 6 %, mais cela est dû en grande partie à la rebudgétisation des crédits de l'ADEME. Par ailleurs, il faut également souligner la baisse d'environ 1,5 % des effectifs affectés à la mission. Je me dois aussi d'évoquer dans le temps qui m'est imparti plusieurs regrets exprimés au sein de la commission. Je commencerai par les territoires à énergie positive pour la croissance verte. Nous le savons tous ici, c'est sur les territoires que la transition se fait aujourd'hui. De nombreuses initiatives ont été prises en matière d'efficacité énergétique, d'économie circulaire et de mobilité. Des promesses ont été faites aux élus pour les encourager dans ces initiatives ; elles ne peuvent être remises en cause par des arbitrages administratifs. les engagements pris doivent être tenus. Le Gouvernement a promis l'inscription de 75 millions d'euros dans le collectif de fin d'année. C'est une première ouverture, mais il faudra aller au-delà. J'espère que vous pourrez nous donner quelques éléments en ce sens. Un autre sujet important est le Fonds chaleur. La promesse présidentielle d'un doublement de ce fonds n'a pas été tenue, alors qu'il s'agit d'un formidable levier pour la production de chaleur à partir de ressources renouvelables ou de récupération.

l'État augmente à un niveau sans précédent les prélèvements sur leurs ressources. Cela n'est pas cohérent et surtout ne peut être durable. Il faudra prévoir de mettre à l'avenir un peu d'ordre dans les ressources des agences de l'eau et les divers prélèvements qu'elles subissent depuis plusieurs années.

Or, nous le savons tous, la sûreté nucléaire est une mission hautement prioritaire de l'État et les dépenses qui lui sont liées vont s'accroître de manière inéluctable au cours des prochaines années.

je commencerai cette intervention par quelques mots sur la méthode. Alors que le changement climatique nous appelle à un changement de paradigme, la représentation nationale dispose d'une petite heure de débat pour examiner les crédits d'une mission fondamentale qui regroupe à elle seule huit programmes, un budget annexe et trois comptes d'affectation spéciale. Comment aborder des sujets aussi vastes que la prévention des risques, les transports maritimes, aériens, fluviaux et ferroviaires, la transition énergétique, le climat, la biodiversité en six minutes ? C'est impossible Je le regrette d'autant plus que, bien qu'en hausse, cette mission est en trompe-l'oeil. Alors qu'elle est censée traduire les engagements du plan Climat, nous n'y retrouvons que très peu de choses nouvelles : il s'agit principalement de revoir les questions du bonus-malus et de la fiscalité sur le diesel. Pour le reste, ce budget se situe dans la continuité des précédents, à une exception notable. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique a été largement réduit à l'Assemblée nationale.

Ainsi, d'après Réseau action climat, l'ensemble des niches fiscales destinées aux énergies fossiles dans les transports représente 7 milliards d'euros annuels. Pourquoi ne pas réorienter cette dépense d'argent public vers une dépense utile pour le climat, nous plaçant ainsi dans un cercle vertueux ? Les personnels du ministère participent à l'effort de réduction de la dépense publique : 828 équivalents temps plein seront supprimés. Or nous estimons, au regard de l'importance de cette mission, que l'emploi public devrait plutôt y être sanctuarisé. N'ayant que peu de temps, et comme nous reviendrons dans nos amendements sur la question spécifique de l'eau et de la biodiversité, je concentrerai mon propos sur la question ferroviaire, qui représente la dépense principale de cette mission. Le rail constitue un levier puissant pour limiter l'émission des gaz à effet de serre. L'état des lieux n'est pas satisfaisant. La part du fret ferroviaire dans le transport de marchandises régresse chaque année faute de soutien des pouvoirs publics, loin des objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement. Cette part n'a eu de cesse de baisser, passant de 24 % en 1990 à 9,6 % en 2017. Or le rail souffre d'une concurrence déloyale de la route, qui bénéficie d'un régime fiscal et social favorable. La dépense fiscale est incontrôlée puisque, pour le remboursement d'une fraction de la TIPP aux routiers, nous passons d'un coût de 400 millions en 2016 à un coût estimé de 1,137 600 millions d'euros supplémentaires pour le transport routier, qui ne participe toujours pas au financement des infrastructures. Pour nous, la question d'une écotaxe reste donc d'une brûlante actualité, au moment même où une révision de la directive Eurovignette est annoncée. les trop rares crédits affectés au fret ferroviaire, notamment dans la loi de finances pour 2017, ont fait partie des crédits annulés. Seuls 90 millions d'euros ont été exécutés pour 2017 sur les 226 millions d'euros prévus. Comment comprendre cette politique alors que l'exigence alors que l'exigence du report modal est incontournable pour respecter nos engagements internationaux sur le climat, et notamment l'accord de Paris ? Au lieu de rendre attractif le rail, ce gouvernement continue de mener une politique de sous-financement qui condamne ce mode de transport face aux Concernant le transport de voyageurs, un projet de loi d'orientation sur les mobilités est attendu au premier semestre de 2018, de même que des scénarios sont à l'étude concernant l'ouverture à la concurrence des transports nationaux de voyageurs. Nous sommes extrêmement inquiets de ces annonces qui sont le prélude d'un nouveau recul du rail. Cette modification de l'organisation des transports fait peser des risques sur la sécurité et la fiabilité des transports, sur un aménagement du territoire qui garantisse le droit de tous à la mobilité. Les lignes non rentables risquent ainsi d'être abandonnées par les nouveaux opérateurs, tandis que SNCF Mobilités s'enferrera dans des difficultés plus grandes encore. Madame la ministre, dans une interview donnée au journal, vous avez déclaré que « les compagnies aériennes, le covoiturage, les cars Macron modifient le champ de pertinence du rail ces déclarations ne sont pas acceptables quand on évalue ces modes de transport sous le prisme de leur bilan carbone. Je rappelle d'ailleurs que nous avions dénoncé à l'époque l'arrivée des bus dits « Macron », comme élément déstabilisant pour les TER et les trains d'équilibre du territoire, dont l'État se débarrasse aujourd'hui sur les régions.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » recouvrent un ensemble de programmes au périmètre très large. Je m'associe

allégeant la charge de cette agence, mais les risques continuent de peser. Les assises nationales de la mobilité, que vous conduisez, madame la ministre, seront donc importantes pour fixer le cap ; notre groupe y sera attentif.

doit nous inviter à engager un grand mouvement de modernisation et de rénovation de ce mode de transport ; Dieu sait qu'il y a à faire ... Cette initiative sera particulièrement importante pour le secteur du fret ferroviaire : l'établissement Fret SNCF est endetté à une hauteur abyssale, et souffre de surcoûts critiques liés à l'organisation du temps de travail. Le Gouvernement doit proposer rapidement des mesures pour anticiper ces changements. du programme 205 « Affaires maritimes », le Gouvernement propose de faire de la sécurité maritime une priorité stratégique. Dans un monde bouleversé par la piraterie, le terrorisme, les migrations de populations et les phénomènes climatiques, la défense de nos mers, en lien, évidemment, avec

Par ailleurs, notre groupe tient à souligner l'importance des crédits accordés à la préservation de l'environnement marin. Le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes porte aujourd'hui une quarantaine d'actions en mer, pour assurer, entre autres, la surveillance des espaces marins protégés, le contrôle des pêches

En écho au débat de notre dernière semaine de contrôle consacré aux énergies de demain, permettez-moi d'évoquer à nouveau la question des énergies marines renouvelables. J'y suis, évidemment, très favorable. Le sujet mérite une grande attention : ce sont des énergies prometteuses, à tous les égards, pour le succès de la révolution énergétique, mais- cela n'est pas rien -elles ne rencontrent pas toujours l'aval des populations locales. Vous connaissez, madame la ministre, mes attaches picardes ; je veux appeler à cet égard toute votre attention sur le risque sérieux que court le projet du Tréport. Ne nous exonérons pas de l'avis des territoires ; nous n'avons pas besoin d'une crise supplémentaire

Le maintien d'un prix unique pour les consommateurs des zones non interconnectées est une bonne chose, et notre groupe sera attentif à sa pérennisation. Quant à la montée en charge des tarifs sociaux de l'énergie, s'il nous semble important de mener rapidement une discussion sur le déséquilibre des traitements entre les énergies choisies, le groupe Les Indépendants - République et Territoires s'engage à préserver ces dispositifs de soutien aux 3 millions de ménages souffrant aujourd'hui des prix de l'énergie. En ce moment, 5 millions de ménages français souffrent non seulement de la faim, mais encore du froid. Ces aides sont essentielles pour protéger les Français. L'État a donc toute sa place à la tête de ces engagements et la généralisation du chèque énergie, expérimenté dans quatre départements depuis mai 2016, nous paraît être une mesure nécessaire dans l'accompagnement des ménages modestes ; il faudra que nous prenions connaissance du rapport sur ces expérimentations. Il faut d'ailleurs que ces ménages soient entendus, c'est la raison pour laquelle nous saluons la dotation de nouveaux moyens en faveur du Médiateur national de l'énergie, dont les compétences ont été élargies par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Sur les programmes 181 et 217, les programmes 181 et 217, représentant ensemble un tiers du budget de la mission, le Gouvernement propose une priorisation des actions avec, néanmoins, des moyens contraints. Notre groupe s'inquiète de la réduction des moyens de l'ADEME, étant donné l'ampleur des tâches à accomplir pour atteindre nos objectifs en matière de transition concerne les programmes 113, 159 et 174, regroupant 10 % des crédits de la mission, il convient de noter que ces budgets doivent prendre en compte la création de la nouvelle Agence française pour la biodiversité. En tant que membre du conseil d'administration de cette agence, je suis son premier budget avec une vigilance quasi affective.

introduite par cet amendement était supprimée par l'Assemblée nationale, l'équilibre financier des politiques de biodiversité en serait menacé. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Gouvernement propose un budget en transition sur ces questions. Nous voterons donc en faveur des crédits de cette mission, mais nous resterons vigilants.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les crédits que nous examinons ce jour doivent être envisagés au travers d'une double optique. La première est celle du court terme, de l'immédiat, de l'instant. C'est l'optique dominante de notre univers, tant les difficultés rencontrées par nos concitoyens sont aujourd'hui nombreuses : difficultés à trouver un emploi ou à le garder, revenus souvent trop modestes, risques pesant sur la qualité de vie en raison d'un environnement dégradé, besoins de mobilité pour travailler ou pour les loisirs ; autant de briques de lien social qui apparaissent immédiatement de manière aiguë dans tous nos territoires. Cette optique dicte aujourd'hui sa loi, et c'est normal, tant les souffrances du quotidien sont immédiatement palpables

pour faire entrer notre pays et ses territoires dans le XXI siècle, il faut avoir un oeil sur le volant et l'autre sur la route et sur l'horizon. Réinventer le modèle français et entraîner notre pays dans la transition écologique et solidaire, c'est bien cette volonté qui sous-tend la dynamique budgétaire du premier projet de loi de finances du quinquennat, que nous examinons ce jour. Les crédits du ministère de la transition écologique et solidaire traduisent concrètement le plan Climat présenté en juillet dernier. Ce plan vise à protéger les plus fragiles, qui sont les premières victimes des dégâts causés par le modèle de développement économique dont nous cherchons à sortir progressivement. Il constitue un objectif transversal, qui se traduit dans l'ensemble des politiques du ministère : l'énergie, les transports, la prévention des risques ou encore la gestion des milieux naturels. Vous me permettrez de citer quelques mesures précisant ces objectifs : le plan de rénovation thermique et le recentrage du crédit d'impôt pour la transition énergétique, la prime à la conversion des véhicules et le soutien aux véhicules électriques, ou encore la croissance du financement des énergies renouvelables, dans le cadre de l'élaboration de la prochaine programmation pluriannuelle pour l'énergie et du grand plan d'investissement voulu par le Président de la République et le Premier ministre. Ce sont autant de traductions concrètes et robustes de l'engagement du Gouvernement en faveur de la préservation du climat et de la planète que l'on retrouve dans ce projet de loi de finances. Ce budget vise également à accompagner et à protéger les plus fragiles. Tel est l'objet du « paquet de solidarité climatique », et en particulier de la généralisation du chèque énergie. C'est aussi en menant conjointement une action résolue dans le domaine de la santé, de l'environnement, de la protection de la biodiversité et de la prévention des risques que nous assurerons cette protection des plus fragiles. En matière de transports, cela a été dit et répété, madame la ministre, il s'agit d'un budget de transition qui marque une nouvelle étape de la réorientation engagée en faveur des transports du quotidien et de la remise à niveau, tant attendue, des réseaux existants. À ce titre, les assises de la mobilité permettront de préparer la loi d'orientation sur les mobilités à laquelle sera associée une loi de programmation équilibrée en ressources et en dépenses. Nous aurons donc l'occasion de débattre largement de ce sujet au printemps prochain. Ce budget clarifie aussi les priorités et dessine le cadre d'action des cinq prochaines années. Non, tout n'a pas été possible dès cette première année, mais, le ministre d'État Nicolas Hulot l'indiquait devant le Conseil économique, social et environnemental mardi dernier, le temps de la concertation est sans doute du temps gagné dans l'action. Le cap est désormais clair et nul doute que ce budget, accompagné du grand plan d'investissement, exprime l'ambition du Président de la République et du Gouvernement pour mettre en oeuvre les feuilles de route données par le Premier ministre au ministre d'État Nicolas Hulot, à vous, madame la ministre, et à vos collègues Brune Poirson et Sébastien Lecornu. Avant de terminer mon intervention, je souhaite insister, au sein de cet hémicycle, sur trois thématiques qui illustrent, je pense, l'ambition forte de ce premier budget, conforme aux engagements du Président de la République. Tout d'abord, sur la mobilité, conformément aux priorités définies par le Gouvernement, les investissements dans le domaine des transports privilégieront les transports de la vie quotidienne, la recherche d'une meilleure efficacité dans l'exploitation des réseaux existants et leur optimisation. Le projet de budget pour 2018 acte le retour d'un État stratège en la matière, un État qui assume enfin pleinement ses responsabilités. N'ayons pas peur de le dire, mes chers collègues, au cours des dernières années, les financements indispensables pour maintenir et régénérer les réseaux existants ont été négligés. La précédente majorité s'était engagée sur de nouveaux projets par trop déconnectés, hélas, des ressources disponibles. Cette situation a conduit à une impasse budgétaire de près de 10 milliards d'euros. Elle a affaibli la parole de l'État, alors que les acteurs ont justement besoin de clarté, de financements lisibles et d'une programmation pluriannuelle de qualité. Sans un cadre précis, il ne nous sera pas possible de tenir nos objectifs de report modal et de modernisation des infrastructures. C'est pourquoi je salue le réexamen du périmètre et des modalités du financement des transports mené au travers des assises nationales de la mobilité lancées en septembre dernier et qui associent l'ensemble des acteurs du territoire pour, notamment, identifier les besoins de chacun et les attentes prioritaires de tous. La politique des transports va désormais s'appuyer pleinement sur les nouveaux usages, en fixant une stratégie claire des mobilités. Elle hiérarchisera mieux les choix d'investissement de la part tant de l'État que des collectivités territoriales. Chers collègues, le budget pour 2018 assainit les bases à partir desquelles le Parlement pourra opérer les choix de financement pluriannuel. D'ores et déjà, nous constatons que la sincérité et la lisibilité du budget sont au rendez-vous. De même, la diminution du taux de la réserve de précaution apporte des marges de manoeuvre inédites, car les gels pénalisaient particulièrement notre programme et l'exposaient aux annulations en cours d'exercice. Loin de marquer un désengagement de l'État, les crédits budgétaires du programme 203 atteindront un montant significatif, en hausse de 200 millions d'euros par rapport à la prévision d'exécution de l'année 2017. Parallèlement, cela a été indiqué, le budget de l'AFITF, porté à 2,4 milliards d'euros, sera également en hausse de 200 millions d'euros, grâce aux recettes fiscales que lui affecte ce projet de loi de finances. Cet effort est prioritairement orienté vers l'entretien et la régénération du réseau national routier non concédé et des canaux. Les concours à SNCF Réseau permettront aussi d'améliorer la rénovation des réseaux existants et de moderniser les systèmes d'exploitation du trafic ferroviaire.

Ces crédits pour 2018 sont donc l'illustration d'un gouvernement résolu à faire rimer long terme et court terme ; voilà pourquoi les sénateurs du groupe La République En Marche le soutiendront. La Monsieur le président, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, comme nous disposons de peu de temps pour étudier ces sujets importants- cela a été dit -, mon intervention se concentrera sur les crédits affectés au financement du transport dans la mission « Écologie, même s'il faut considérer que les mobilités sont transversales et entrent en ligne de compte dans le plan Climat, dans les enjeux de santé publique, dans la politique de la ville ou encore dans le développement économique. La présentation budgétaire de ces crédits en dit long sur la situation des transports dans notre pays, alors que tout le monde en reconnaît l'importance pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Une part seulement de ces crédits est retracée en loi de finances, et encore de façon éclatée, puisqu'ils sont répartis entre le programme 203 « Infrastructures et services de transport », les deux comptes d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Enfin, une part des crédits des transports, composée des taxes affectées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, l'AFITF, ne figure pas dans le projet de loi de finances, un collègue

la ministre. Cet éclatement et ce manque de visibilité budgétaire sont symptomatiques de la difficulté que nous avons à mettre en place une vraie politique des transports qui obéisse à un plan d'ensemble. C'est bien ce que nous attendons des assises de la mobilité qui se sont ouvertes en septembre dernier, sous votre présidence, madame la ministre, et dont les conclusions serviront de base au projet de loi d'orientation sur les mobilités. J'ai eu personnellement l'occasion de participer au lancement de ces

L'État a pris trop d'engagements, ce qui a conduit le Gouvernement à décréter une pause dans les grands projets d'infrastructures, alors que les citoyens sont en attente. C'est à la faveur de cette pause que le budget de 2,4 milliards d'euros, prévu pour l'AFITF, pourrait sembler suffisant. la situation financière de cet établissement n'en demeure pas moins préoccupante. Comme l'ont rappelé nos rapporteurs, dont je salue au passage l'excellent travail, l'AFITF aura à débourser 12,3 milliards d'euros dans les années à venir à venir ; nous n'en avons pas fini de payer le camouflet de l'écotaxe ... La dette de SNCF Réseau compromet également son action de modernisation du réseau ferré. On ne peut que s'inquiéter de voir notre rapporteur remettre en cause la crédibilité du contrat de performance décennal signé entre cet établissement et l'État. La non-soutenabilité caractérise également le financement du Grand Paris Express, dont le coût, initialement évalué à 25 milliards d'euros, déraperait pour atteindre la bagatelle de 35 milliards d'euros ! Voies navigables de France va de son côté devoir mettre en oeuvre un plan social du fait de l'obsolescence de la taxe hydraulique. Il n'y a guère que le secteur de l'aviation qui se maintienne, cela a été évoqué, malgré la forte concurrence internationale. Il faut donc rester vigilant sur ce sujet.

Nous ne pouvons par exemple que soutenir l'effort de 200 millions d'euros consenti en direction de l'AFITF pour rénover les réseaux existants et améliorer les transports du quotidien. Pour toutes ces raisons, et sous réserve des réformes de structure à venir, le groupe Union Centriste soutiendra les crédits transport de cette mission. Très bien

Monsieur le président, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, voilà un peu plus d'un an, le 4 novembre 2016, la diplomatie française remportait un succès inégalé sur le terrain de la lutte contre le réchauffement climatique, en obtenant la ratification de l'accord de Paris par 55 États représentant représentant 55 % des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 168 États cumulant plus de 80 % des émissions de gaz à effet de serre qui l'ont ratifié. Le changement climatique devient une réalité palpable pour chacun de nous. Prenons un exemple simple, l'extinction, en Europe, des insectes pollinisateurs, comme les abeilles ou les papillons. Des études très sérieuses démontrent combien nos écosystèmes sont en danger, certaines atteintes étant même irréversibles. Eh oui ! Il est donc urgent d'agir, d'autant plus que la COP23 s'achève sans grand engagement, excepté pour ce qui concerne le charbon. L'avertissement lancé par 15 000 scientifiques, le 13 novembre dernier, contre la mutilation définitive infligée à notre planète ne doit pourtant pas demeurer lettre morte À bien des égards, ce budget de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » s'inscrit dans la continuité des budgets précédents, ... C'est vrai ! ... et affiche sa volonté d'accélérer la transition énergétique. Vous présentez ce budget comme la mise en musique du plan Climat, ce fameux annoncé en juillet dernier : recentrage du crédit d'impôt, généralisation du chèque énergie, extension de la prime à la conversion des véhicules polluants avec doublement de la prime de 1 000 euros pour les ménages à revenus modestes, ou encore hausse de la fiscalité énergétique, au travers de la taxe carbone.

C'est un outil unique de gouvernance, qui peut nous permettre d'affronter les défis du changement climatique et de la sixième extinction de masse provoquée par l'homme. En revanche, nous nous interrogeons fortement sur la pérennité du financement des agences de l'eau,

ainsi que le prélèvement, en 2018, de 200 millions d'euros sur leur fonds de roulement. Beaucoup de parlementaires, dont ceux du groupe socialiste et républicain, se sont opposés à cette baisse de plafond et, si le Sénat en a acté la suppression, celle-ci sera très certainement remise en cause par l'Assemblée nationale.

de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS, pour un montant compris entre 30 millions et 37 millions d'euros. Cet article suscite également des questions. L'étude d'impact de ce projet de loi reconnaît ainsi que, si cette mesure est neutre pour les organismes visés- AFB

les industriels et enfin les particuliers. Attention à ne pas bousculer les équilibres en place ! En outre, en ce qui concerne le financement de l'ONCFS, qui constitue un vrai coût supplémentaire pour les agences de l'eau, l'étude d'impact précise que « cette mesure devrait inciter les agences de l'eau à prioriser leurs dépenses, à travers la rationalisation de dispositifs d'intervention dont l'efficience et l'efficacité n'ont pas été démontrées Vous pouvez comprendre, madame la ministre, que cette seule déclaration suscite des interrogations de notre part et qu'elle nécessite des précisions. Je ne reviendrai pas sur nos craintes concernant les territoires à énergie positive, Roland Courteau s'en chargera dans quelques instants. Je souhaite plutôt aborder

structure à laquelle je suis particulièrement attaché en tant qu'élu des Ponts-de-Cé, dans le Maine-et-Loire, où siège le CEREMA Ouest. Cette diminution, même si elle est légèrement compensée par une augmentation de ses ressources propres, nous inquiète fortement, car elle est combinée à une forte diminution des emplois. En effet, le CEREMA est un interlocuteur essentiel des collectivités territoriales en matière d'ingénierie et de conseil. Espérons que la future agence nationale de la cohésion des territoires saura préserver les missions et les effectifs de cette structure, qui accompagne efficacement les collectivités dans leurs projets environnementaux. transports » de la mission, nous savons qu'il s'agit là d'un budget de transition, dans l'attente des résultats des assises de la mobilité. La remise à plat des investissements destinée à reprioriser les grands projets de transports sur le territoire va dans le bon sens. très attentifs aux propositions formulées en début d'année prochaine par le Conseil d'orientation des infrastructures. Un autre dossier retiendra notre attention pour l'année 2018, je veux bien sûr parler de l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire, qui devra garantir le bon accomplissement des missions de service public.

Je me permettrai donc, madame la ministre, d'exprimer quelques interrogations, et j'écouterai évidemment avec attention vos réponses précises. La première interrogation concerne les moyens humains du ministère. Vous prévoyez, cette année encore, une baisse sensible des moyens humains consacrés à l'écologie. Pourtant, sans fonctionnaires- je crois que nous en serons tous d'accord, et c'est l'occasion de leur rendre hommage -, aucune politique publique ne peut être mise en oeuvre.

En complément de cette inquiétude, j'ai deux autres interrogations portant sur les budgets de ces agences essentielles que sont l'Agence française de la biodiversité et l'ADEME. Pour ce

Parmi les plafonnements discutables, nous dénonçons aussi le plafonnement de la ressource affectée au Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Vu les enjeux, notamment le risque d'inondation et de submersion marine,

Monsieur le président, madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je souhaite remercier tout d'abord l'ensemble de mes collègues, les rapporteurs et le Gouvernement pour le travail réalisé dans le cadre de l'examen de ce texte. La mission « Écologie, développement et mobilités durables » est composée de huit programmes, cela a été dit à plusieurs reprises. Les sujets concernés par ces derniers revêtent tous d'une importance particulière pour notre pays : transition énergétique, climat, biodiversité, mobilité, énergie, entre autres. Les crédits de la mission sont en hausse pour l'exercice 2018, avec 11,35 milliards d'euros d'autorisations d'engagement contre 10,2 milliards d'euros en 2017. Cette augmentation permet simplement à la France de garder un minimum de cohérence avec ses engagements nationaux et internationaux. C'est un budget qui, après examen approfondi, manque clairement de souffle pour inspirer une politique volontariste sur ces sujets essentiels. J'ai la conviction que ces enjeux méritent davantage de considération. Cela étant dit, il me serait impossible d'aborder les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » sans évoquer la première partie du projet de loi de finances. Aussi, permettez-moi de revenir sur la vision politique du Gouvernement concernant ces nombreux sujets, à travers l'examen des crédits. Pour le secteur des transports, qui est le secteur émettant le plus de gaz à effet de serre en France, à savoir près de 30 % de la totalité des émissions, les mesures concernant le renforcement de la prime à la conversion automobile et son élargissement sont à saluer. Je reviendrai sur le transport tout à l'heure. Deux sujets de cette mission doivent mobiliser toute notre attention, car ils seront au coeur des discussions de la commission mixte paritaire. Il s'agit du budget des agences de l'eau et du Fonds de prévention des risques naturels majeurs.

à hauteur de 2,105 milliards d'euros. L'Assemblée nationale a voté un amendement du Gouvernement rectifiant ce plafond, mais en instaurant, en contrepartie, un prélèvement de 200 millions d'euros sur la trésorerie des agences.

Prenons comme exemple l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Ces prélèvements aboutiraient à ramener la trésorerie de l'agence à 4 millions d'euros et à des reports de paiement de subventions sur 2019. En résumé, ce prélèvement de trésorerie met en difficulté l'ensemble des acteurs de la chaîne, des agences de l'eau jusqu'aux collectivités qui investissent. Le Sénat a adopté une position de compromis et n'a pas supprimé ce prélèvement. J'invite donc le Gouvernement à être particulièrement attentif- nous le serons pour ce qui nous concerne -sur l'évolution financière des agences de l'eau et sur leur capacité à remplir pleinement leur rôle. Le second sujet de préoccupation que je souhaite aborder concerne le fonds de prévention des risques naturels majeurs, évoqué à l'instant par mon collègue Ronan Dantec. Je me permets de rappeler que ce fonds, dit dit fonds Barnier, est entièrement alimenté par un prélèvement sur les primes des bénéficiaires d'un contrat d'assurance habitation ou véhicule au titre de la garantie catastrophe naturelle, c'est-à-dire par l'ensemble des citoyens, des associations, des collectivités et des entreprises. Le Gouvernement prévoyait de plafonner ce fonds dans la limite de 137 millions d'euros, alors que les recettes, en 2018, devraient s'élever à 208 millions d'euros- au passage 71 millions d'euros de trésorerie prélevés pour le budget, après 55 millions d'euros en 2016 et un peu plus en 2017. Ce projet a logiquement soulevé l'incompréhension sur toutes les travées du Sénat. En effet, comment imaginer plafonner pour la première fois ce fonds au regard des récentes catastrophes climatiques qui ont touché notre pays ! Comment, quelques mois après le terrible ouragan Irma, peut-on défendre l'idée de priver ce fonds des moyens nécessaires pour honorer ses engagements ? Je remercie sur ce sujet l'ensemble de mes collègues, qui ont largement voté l'amendement de suppression de ce plafonnement que j'avais déposé, de la même façon que mon collègue Ronan Dantec. J'invite le Gouvernement et l'Assemblée nationale à suivre cette décision dans le cadre des discussions à venir. De nombreux points restent cependant en suspens, cela a été évoqué également à plusieurs reprises. Je pense aux contrats conclus par 500 collectivités dans le cadre du plan Territoire à énergie positive pour la croissance verte.

La dégradation de la qualité de notre réseau routier doit également être soulignée. Les crédits sont en augmentation de 100 millions d'euros, malgré tout, pour atteindre 802 millions d'euros pour 2018. Cependant, un audit interne du ministère des transports estime, pour sa part, qu'il faudrait 1 milliard d'euros chaque année jusqu'en 2027 pour remettre réellement l'ensemble du réseau routier à niveau. J'évoquais, au début de mon intervention, un budget qui manque de souffle. Cette expression s'applique parfaitement aux crédits du programme 205 « Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture Je remercie à ce titre mon collègue Charles Revet qui, dans son rapport pour avis présenté par Michel Vaspart, met en exergue cette absence totale de vision politique pour l'économie maritime, tout cela un an après la loi Leroy. En effet, seuls 240 millions d'euros devraient être consacrés à la politique maritime. Ces fonds sont largement insuffisants.

nécessaire à l'intermodalité entre autres, Voies navigables de France a rappelé qu'un investissement de 100 millions d'euros par an pendant dix ans serait nécessaire pour sécuriser et régénérer l'ensemble des aménagements fluviaux afin d'encourager ce moyen de transport vertueux. Pour terminer sur ce sujet, permettez-moi de rappeler la volonté initiale du Gouvernement, ou de Bercy, de supprimer l'exonération des charges sociales en faveur des entreprises d'armement maritime battant pavillon français pour leur personnel embarqué, pourtant votée dans la loi pour l'économie bleue de 2016. L'article

Je ne peux que déplorer le manque de financements en faveur de l'économie maritime qui, je le rappelle, est l'équivalent de l'aéronautique ou de l'automobile en France, soit 14 % du PIB, 270 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en intégrant l'ensemble des activités. J'aurais pu citer le budget de l'ADEME, le Fonds chaleur, la politique des déchets, le fret ferroviaire, le CEREMA, mais il n'est pas possible de détailler l'ensemble des actions des huit programmes de cette mission. Pour conclure, le budget de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » est un budget sans véritable relief ou réelles perspectives.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à la suite des propos de Joël Bigot, une chose est certaine le XXI siècle ne saurait être la répétition du précédent, au cours duquel la consommation d'énergie a été multipliée par deux, avec abondance de gaz à effet de serre et d'atteintes à la biodiversité. Aujourd'hui, nous devons faire face à des défis climatiques et environnementaux, et c'est là une grande cause et c'est là une grande cause nationale, européenne et planétaire. Pour la première fois en effet, l'humanité est en mesure d'anéantir sa propre espèce. La politique énergétique actuelle s'inscrit donc, et c'est bien ainsi, dans la continuité de celle qui a été impulsée par les précédents gouvernements. dommage que certains manques viennent gâter quelque peu cette politique énergétique ; j'y reviendrai. Quelques simples remarques auparavant, car le temps m'est compté. Concernant les dépenses fiscales,

nous ne pouvons en revanche approuver les restrictions apportées sur les chaudières à fioul à haute performance ou sur les fenêtres. Par rapport aux certificats d'économies d'énergie, nous aurions apprécié de disposer d'une évaluation de leurs performances auprès, notamment, des ménages les plus précaires. De plus, et face à l'arnaque dont ils font l'objet, il serait temps que le Pôle national des certificats d'économies d'énergie puisse disposer d'un service de contrôle qui ne soit pas sous-dimensionné face à l'immensité de sa tâche. Concernant le chèque énergie, nous considérons que l'on serait bien inspiré d'en relever non seulement le seuil d'éligibilité, qui nous paraît être vraiment trop bas par rapport au seuil de pauvreté, mais également le montant. Par rapport à l'augmentation de la fiscalité dans le cadre de la stratégie nationale attention aux conséquences d'une fiscalité lourde sur les ménages de condition modeste. Son impact est loin d'être anodin. Nous défendrons un amendement amendement visant à accompagner les primes à la conversion de la mise en place de prêts à taux zéro. Enfin, j'en arrive au désengagement de l'État et au durcissement des règles de gestion des conventions relatives aux 500 lauréats des TEPCV.

Avec Franck Montaugé et mes collègues, je défendrai un amendement visant à abonder le fonds de financement : la transition se fera avec les territoires ou ne se fera pas. Autre question, madame la ministre : où en est-on du doublement du Fonds chaleur ? Enfin, je souhaite attirer votre attention sur la très forte consommation d'électricité liée à l'essor de l'écomobilité dans les prochaines années. Comment nos réseaux de transport et de distribution d'électricité vont-ils pouvoir répondre à cette forte demande et, en même temps, à l'arrivée massive des énergies renouvelables

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le périmètre de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » et des comptes spéciaux associés est si vaste qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de porter un avis détaillé sur l'ensemble des crédits dans le temps imparti. Mon intervention portera donc simplement sur deux points qui ont suscité des débats animés au sein de notre assemblée lors du vote de la première partie du projet de loi de finances et encore cet après-midi. Je commencerai par la fiscalité sur l'eau. aquatiques, l'ONEMA, à hauteur de 108 millions d'euros, puis de 145 millions d'euros, par un prélèvement sur les taxes fiscales perçues par les agences de l'eau auprès des usagers de l'eau, pouvait se comprendre puisque cet organisme, créé en 2007, venait appuyer les services de l'État et ceux des agences de l'eau pour mettre en oeuvre la politique de l'eau. Les deux principes fondamentaux de la politique de l'eau- « l'eau paie l'eau » et « pollueur-payeur »-étaient respectés. la biodiversité, l'AFB, en 2017, avec la fusion de l'ONEMA dans la nouvelle structure, et l'extension du périmètre d'intervention des agences de l'eau à la biodiversité terrestre et marine, deux propositions inscrites dans la loi sur la biodiversité de 2016, ont constitué une rupture. C'était la première étape d'un financement de la biodiversité par les usagers de l'eau et, en premier lieu, par les consommateurs d'eau potable qui acquittent plus de 80 % des taxes perçues par les agences de l'eau. Le budget 2018 marque une nouvelle rupture : le Gouvernement a choisi de faire financer par les agences de l'eau, et donc par les usagers et les consommateurs d'eau, les subventions pour charges de service public qui étaient antérieurement versées à partir du budget de l'État aux organismes intégrés dans l'AFB. Cela peut s'entendre pour ce qui concerne l'ex-Agence des aires marines protégées, si l'on considère qu'il existe une continuité entre les eaux continentales et les eaux marines. comment justifier que les subventions pour charges de service public versées à l'ONCFS et aux parcs nationaux, deux établissements publics qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'eau, soient dorénavant financées par les agences de l'eau ? À l'évidence, il n'y a pas d'autre justification que la débudgétisation. Cette décision marque un changement profond de philosophie dans la fiscalité de l'eau. En effet, la loi sur l'eau de 1964 a donné naissance aux premières taxes à visée environnementale, bien avant que l'on parle de fiscalité écologique. Ces taxes, telles qu'instituées par le législateur, avaient vocation à financer les agences de l'eau, charge à ces dernières de soutenir des actions permettant aux industriels, aux agriculteurs, aux collectivités de préserver la ressource en eau. Cette philosophie a été confortée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 qui a donné un pouvoir de contrôle au Parlement sur ces taxes, ainsi que sur leur utilisation. Elle est aujourd'hui remise en cause. La débudgétisation prévue par le projet de loi de finances pour 2018 transforme ces taxes en un impôt de rendement. L'eau devient une assiette fiscale ordinaire, ce qui est contraire à la volonté constante du législateur. Si l'on veut faire financer la biodiversité par les agences de l'eau, il faut mettre en cohérence l'origine de leurs recettes avec la nature de leurs dépenses. En application du principe « pollueur-payeur », il faut diversifier les assiettes contributives et mettre à la charge des activités qui dégradent la biodiversité terrestre le financement des mesures qui assurent sa protection et sa restauration. Voilà un chantier concret de fiscalité écologique pour éviter de faire du consommateur d'eau une simple vache à lait. Nous invitons le Gouvernement à nous faire des propositions concrètes en ce sens pour les prochaines lois de finances. Dans un autre domaine, la fiscalité sur les produits énergétiques pose également question. La forte hausse de la contribution climat-énergie décidée par votre gouvernement,

En effet, une taxe carbone de 10 euros par tonne de CO2 induit des recettes de TICPE de 2,3 milliards d'euros, qui se montent à près de 3 milliards d'euros en tenant compte des recettes de TVA. Nous ne nions pas le rôle incitatif que peut jouer une fiscalité punitive sur la consommation de ressources énergétiques. Nous pensons cependant que les recettes de cette fiscalité doivent être fléchées vers des actions en faveur d'une modification des comportements, d'une mitigation des nuisances sur l'environnement. Dans le budget 2018, le compte n'y est pas La croissance de 3,7 milliards d'euros des recettes de TICPE se traduit seulement par une augmentation de 100 millions d'euros de l'enveloppe de la prime à la conversion et de 80 millions d'euros des crédits alloués au chèque énergie qui s'est substitué aux tarifs sociaux. Le gain net pour l'État est donc de 3,5 milliards 3 milliards d'euros, soit le montant des exonérations de taxe d'habitation ! Votre gouvernement ne serait pas le premier à utiliser la fiscalité sur les produits énergétiques pour financer d'autres politiques. En 2016, la croissance de la TICPE a largement contribué au financement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Pour autant, les besoins de financement en faveur de l'environnement existent. Déjà en 2016, les sénateurs avaient attiré l'attention du Gouvernement sur le manque de ressources financières des régions et des EPCI pour mettre en oeuvre les schémas environnementaux, dont ils ont désormais la responsabilité,

Le concours financier de l'État est conditionné à la signature d'un contrat d'objectifs. Donner aux collectivités les moyens financiers d'informer et de mobiliser les acteurs locaux, de renforcer la performance énergétique du patrimoine urbain, de développer une mobilité urbaine faiblement émettrice en gaz à effet de serre et de favoriser les énergies renouvelables, voilà des actions concrètes, au plus près du citoyen, qui donneront du sens à la réduction de son pouvoir d'achat. Nous espérons que les députés ne remettront pas en cause la sagesse des sénateurs. Comme l'a dit précédemment Didier Mandelli, le groupe Les Républicains s'abstiendra sur les crédits de la mission.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie pour l'ensemble de vos interventions, d'autant que j'ai noté, mesdames, messieurs les rapporteurs,

je voudrais préciser en quelques mots l'esprit dans lequel ce budget a été construit. Le budget, vous le savez, est la clé de voûte de l'action politique. Il exprime les ambitions que porte le Gouvernement pour répondre au défi de la transition dans laquelle nous plaçons notre action. Il traduit les grands choix que nous faisons pour la transition écologique et solidaire, et les transports. Il repose sur trois principes : un principe de sincérité et de participation équitable au redressement des comptes publics une exigence de continuité des actions engagées pour la transition énergétique et écologique, tant il paraît indispensable de maintenir dans le temps un effort prolongé pour faire face au défi climatique dans toutes ses composantes une recherche de mobilisation de moyens complémentaires pour accompagner cette transition, avec la conviction qu'elle doit également être solidaire. Tout d'abord, le budget du ministère est sincère : il a fallu pour cela consacrer des moyens importants au financement des engagements passés. Le Gouvernement a en effet choisi d'assumer les contraintes budgétaires avec lisibilité et transparence. C'est un exercice difficile, notamment dans le secteur des transports dont j'ai la responsabilité directe, mais il est indispensable. C'est notamment le sens de la pause annoncée par le Président de la République sur nos grands projets : ce n'est pas par plaisir, mais pour permettre de poser des choix en matière d'infrastructures. Je note, à cet égard, l'excellent rapport de votre Haute Assemblée, dont nous pouvons largement nous inspirer pour faire le bilan des choix en termes d'infrastructures. le Parlement aura à en débattre, notamment dans le cadre du projet de loi de programmation des infrastructures, et cela me semble essentiel, car ils sont fondamentaux. en particulier choisir la part allouée à la poursuite des grands projets. Le sénateur Marchand l'a rappelé, nous sommes confrontés à une impasse de 10 milliards

à l'aménagement de nos réseaux, afin de les mettre aux niveaux promis de contrat de plan en contrat de plan. Il s'agit de sortir des promesses non financées et de redonner du crédit à la parole de l'État, et je remercie Mme la sénatrice Keller, ainsi que MM. les sénateurs Corbisez et Cornu, de soutenir cette démarche. Autre exemple de cette exigence de sincérité budgétaire, l'ADEME, qui illustre les difficultés pouvant résulter d'une budgétisation insuffisante de crédits telle qu'on l'a connue encore au cours de l'année 2017. Vous le savez, l'ADEME avait alerté les élus sur ses problèmes de trésorerie. Pour y faire face, elle bénéficiera, en 2018, d'un important recalibrage de ses crédits de paiement, en augmentation de 31 %, ce qui lui permettra de couvrir ses échéances. Cette « remise à flot » de l'ADEME était indispensable, car elle est un acteur majeur pour la mise en oeuvre de la transition écologique et solidaire, avec des interventions importantes pour soutenir les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables, notamment au travers du Fonds chaleur, le développement de l'économie circulaire par l'intermédiaire du Fonds déchets, le soutien à la mobilité durable et l'innovation dans ces différents domaines, ainsi que des interventions pour la mise en sécurité des sols pollués. Le budget du ministère permet en outre de poursuivre et d'accentuer l'effort entrepris pour aller vers une économie décarbonée et solidaire. Dans la continuité de l'accord de Paris et pour renforcer l'action de la France au travers du plan Climat, nous avons engagé la sortie des énergies fossiles, en tout cas pour les véhicules, d'ici à 2040. Nous l'avons fait en prévoyant, dans ce projet de loi de finances, une trajectoire d'augmentation du prix du carbone pour inciter les acteurs à réduire leur consommation d'énergies fossiles. La tonne de CO2, qui sert, je le rappelle, de base au calcul des taxes intérieures de consommation, doit ainsi passer de 30,50 euros en 2017 à 44,60 euros en 2018, pour atteindre progressivement 86,20 euros en 2022. Par ailleurs, nous avons décidé d'accélérer le calendrier de la suppression de l'avantage donné au diesel, qui paraît aujourd'hui totalement injustifié compte tenu de la pollution de l'air par les émissions de particules fines issues de sa combustion ; je sais que c'est un sujet, monsieur le sénateur Husson, auquel vous êtes particulièrement sensible. Le tarif de la TICPE appliqué au gazole se rapprochera de celui appliqué aux essences de façon à annuler progressivement, d'ici à quatre ans, l'avantage fiscal accordé au diesel. Évidemment, l'augmentation de ces prélèvements se place, je voudrais le souligner auprès du sénateur Gremillet, dans le cadre d'une baisse globale des prélèvements obligatoires. C'est donc l'ensemble de ces équilibres qu'il faut regarder,

» repose notamment sur trois mesures. Tout d'abord, la prime à la conversion de véhicules diesel anciens permettra d'accompagner les ménages pour acquérir des véhicules moins polluants, y compris des véhicules d'occasion. Cette mesure devrait permettre le renouvellement de 100 000 véhicules en 2018.

quelle que soit la source d'énergie. C'était bien le problème posé par les tarifs sociaux précédemment. Ce chèque énergie pourra également soutenir des travaux de rénovation énergétique

avant la mise en oeuvre d'une prime à la rénovation énergétique versée à compter de 2019 dès la réalisation des travaux. En complémentarité avec cette politique visant à intégrer dans le prix du carbone le coût de ses externalités négatives, le développement de nouvelles sources d'énergie renouvelable continue à constituer une priorité pour le ministère. Au total, plus de 6,5 milliards d'euros seront consacrés au développement de l'énergie renouvelable.

L'enjeu pour le ministère est bien d'optimiser, notamment dans le cadre d'appels d'offres, l'efficacité des aides en tenant en compte des particularités de ces filières.

Dans nos grandes métropoles, des millions de nos concitoyens sont en effet confrontés à la saturation de leurs réseaux de transport, qu'il s'agisse des routes ou des transports publics. Dans nos territoires ruraux, des millions de personnes se sentent à juste titre isolées, car les investissements nécessaires au désenclavement- une route correcte, une voie ferrée entretenue -n'ont pas été réalisés. La qualité et l'optimisation des réseaux et services existants, ferroviaires, routiers ou fluviaux, sont un préalable nécessaire. Le maintien, voire le renforcement des moyens qui leur sont consacrés par le budget de l'État en 2018 est donc une première traduction de nos priorités.

Par ailleurs, je peux confirmer à M. le sénateur Cornu et à Mme la sénatrice Keller les commandes de l'État pour les trains d'équilibre du territoire seront honorées pour l'ensemble des régions en 2018. Vous le savez, les assises de la mobilité qui s'achèvent vont permettre d'identifier les besoins et les attentes prioritaires des Français en termes de mobilité à l'horizon de 2030, mais aussi de faire émerger de nouvelles solutions. Un projet de loi d'orientation sur les mobilités sera présenté pour être débattu au Parlement au premier semestre de 2018. Pour la première fois, un projet de loi de programmation des infrastructures

et en lien avec la priorité accordée aux réseaux existants, il nous est apparu nécessaire d'augmenter de 200 millions d'euros les recettes de l'AFITF dès 2018.

Vous l'aurez compris, monsieur le président, mesdames messieurs les sénatrices, ce budget traduit dès 2018 les orientations que nous souhaitons prendre tout au long du quinquennat. Je n'aurai certainement pas le temps de répondre à toutes vos questions, mais je voudrais rapidement apporter quelques précisions

dont la cohérence est absolument essentielle, ne sera pas remis en cause. Monsieur le sénateur Capo-Canellas, j'ai bien noté les inquiétudes sur les différents opérateurs que sont Météo France, l'IGN, Pour Météo France, je confirme que le Gouvernement est déterminé à lancer en 2018 l'acquisition du supercalculateur, l'investissement étant inscrit dans la trajectoire budgétaire pluriannuelle. Excellent ! S'agissant de l'IGN, je suis d'accord sur la nécessité de tirer les conséquences de l'Une mission de réflexion sera engagée sur ce sujet au début de l'année prochaine. Le CEREMA, mentionné par plusieurs orateurs,

et de ses agents. Cette mission sera lancée dans les prochains jours et devra être menée en cohérence avec les réflexions en cours sur l'Agence de la cohésion des territoires.

que nous avons lancée sur le secteur ferroviaire et qui devrait aussi trouver une concrétisation très rapidement dans le cadre de la conférence des sillons, qui se tiendra d'ici la fin de l'année. La priorité pour redresser le fret ferroviaire, c'est d'être capable de faire rouler des trains de fret de manière efficace sur le réseau ferré national.

Quant à la privatisation d'Aéroports de Paris, vous savez que cette entreprise a un statut très particulier puisqu'elle est propriétaire de son foncier et des infrastructures qu'elle exploite. C'est évidemment un acteur stratégique de l'accessibilité, non seulement à l'Île-de-France, mais aussi à l'ensemble du territoire national.

qui vise à repenser le rôle de l'État et son mode d'action et à réfléchir au niveau des effectifs dans le cadre d'une réflexion globale.

afin d'assurer l'intégralité du financement des territoires à énergie positive pour la croissance verte prévu par le précédent gouvernement, soit 750 millions d'euros. Une circulaire envoyée le 26 septembre dernier par le ministre de la transition énergétique et solidaire expliquait devoir limiter les crédits de paiement destinés à financer les territoires à énergie positive pour la croissance verte à 400 millions d'euros.

» et à « appliquer strictement » de nouvelles règles de gestion « destinées à recentrer le dispositif » des TEPCV. Ce désengagement de l'État, à hauteur de 350 millions d'euros, et le durcissement des règles de gestion des conventions relatives aux 500 lauréats des TEPCV inquiètent fortement les élus locaux qui se sont engagés dans la transition énergétique. Certes, face à la montée de ces inquiétudes dans les territoires, le Gouvernement s'est voulu rassurant, en assouplissant, d'une part, les règles et critères de sélection des TEPCV et en abondant, d'autre part, en loi de finances rectificative, le programme 174 « Énergie, climat et après-mines » de 75 millions d'euros.

Néanmoins, ces amendements, tels qu'ils sont proposés, auraient pour conséquence d'amputer le programme 159 de plus de 50 % de ses crédits. Serait ainsi supprimée la moitié du budget de Météo France, du CEREMA et de l'IGN, dont nous avons pourtant la situation sensible. Par ailleurs, l'enveloppe spéciale « transition énergétique », qui finance les TEPCV, n'a pas besoin de 275 millions d'euros de crédits supplémentaires en 2018,

des crédits disponible à 250 millions d'euros, soit l'équivalent des besoins de financement au titre de l'année 2018. Les porteurs de projets ont

de même assez surpris. Le Sénat avait pris la décision assez courageuse de rendre obligatoires les plans climat-air-énergie territoriaux sur l'ensemble des territoires, en créant une compétence nouvelle. Or les PCAET ont totalement

dernier : « Vous êtes très nombreux à vous inquiéter des remises en cause budgétaires brutales qui vous ont été notifiées. Je partage votre inquiétude, d'autant que rien ne justifie le fait que l'État ne respecte pas sa signature. En effet, je viens

explication de vote.

qui se termineront le 13 décembre prochain. Je peux vous assurer que l'une des priorités de ces assises est de proposer des solutions alternatives à la voiture individuelle pour les populations- nombreuses

Depuis la loi Oudin-Santini de 2005, les agences de l'eau réalisent, en étroite collaboration avec les collectivités territoriales, des programmes de développement sanitaire indispensables pour les pays émergents dans les domaines de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement, et donc de la santé. En tant que vice-président en charge de la coopération décentralisée à l'agglomération d'Angers, poste que je n'occupe plus, j'ai pu bénéficier de l'expertise essentielle des agences de l'eau en vue de la création de puits permettant l'accès à l'eau potable dans la région de Bamako au Mali. Selon le dernier rapport d'activité des agences de l'eau paru en septembre 2017, la participation à ces programmes de coopération s'élevait à 15 millions d'euros en 2016. Alors que le Président de la République vient d'assister à un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, il semblerait judicieux de ne pas interrompre les programmes de coopération qui fonctionnent particulièrement bien en Afrique de l'Ouest et pour lesquels les besoins sont immenses.

Les agences de l'eau sont doublement touchées. Premièrement, elles participent au budget de l'État à hauteur de 200 millions d'euros cette année. Le « plafond mordant » a, en effet, été repoussé à la discussion budgétaire pour 2019.

Si la participation des agences de l'eau au financement de l'AFB a été actée par la loi sur la biodiversité, le financement de l'ONCFS et des parcs nationaux semble être une nouvelle étape dans le désengagement de l'État. Une étape qui ne respecte pas le principe défini depuis l'adoption de la loi sur l'eau de 1964, qui veut que « l'eau finance l'eau

Les agences de l'eau sont fortement impactées par vos arbitrages budgétaires, madame la ministre. La perte est estimée, par certains acteurs, à 20 % de leur budget, ce qui semble déraisonnable. Pourtant, les missions des agences de l'eau sont fondamentales pour la préservation de la ressource et l'accompagnement des collectivités. plus indispensable que les collectivités doivent prochainement exercer la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, aussi appelée GEMAPI. Ce désengagement de l'État est préjudiciable à la pérennité du financement de l'Agence française pour la biodiversité, de l'ONCFS et des parcs nationaux,

l'allocation d'une partie des recettes des agences de l'eau au financement de la politique de la biodiversité et de la chasse irait totalement à l'encontre

Si, par cet article, le Gouvernement entend faciliter la lecture des moyens consacrés aux opérateurs de la biodiversité,

Le Gouvernement entend maintenir le mécanisme qui renforce le rôle central des agences de l'eau dans le financement de la politique de l'eau et de la biodiversité. Je rappelle que

qu'elles sont un levier considérable au service des politiques de l'eau, de la biodiversité, de la mer, mais aussi de la cohésion des territoires. Je rappelle aussi

lieu sur le niveau nécessaire des ressources de la politique de l'eau. Nous proposons de le faire en deux temps. D'abord, une mission conjointe d'inspection sur les agences de l'eau et les opérateurs de la biodiversité nous permettra d'évaluer si l'organisation est adaptée et si les choix opérés soulèvent des difficultés. Ensuite, nous réunirons des assises de l'eau. Annoncées par le Président de la République lors du congrès des maires, elles permettront

va prochainement s'ouvrir sur le financement de la politique de l'eau, je vous propose de retirer ces amendements ; sinon, l'avis du Gouvernement sera défavorable.

extrêmement important. Enfin, l'augmentation de la population de 50 000 habitants par an va poser des problèmes certains. Nous devons absolument anticiper et prévoir ; c'est notre rôle de politiques. Nous ne pouvons pas faire comme si le réchauffement climatique n'était pas en marche et qu'il n'avait aucun impact sur la ressource en eau. Ne faisons pas comme si nous

Année après année, les ressources des agences de l'eau sont considérées comme une variable d'ajustement du budget général. « Plafond mordant », prélèvement sur le fonds de roulement, financement des autres agences de l'État ... À force de ponctions, les agences ne peuvent plus faire face à leur coeur de mission. Pourtant, ces missions sont essentielles pour la préservation de la ressource et l'accompagnement des acteurs de l'eau. Au moment où l'urgence climatique est posée, où nous avons une conscience collective de plus en plus forte des conséquences des activités humaines sur notre environnement, une telle démarche gouvernementale apparaît incompréhensible.

Comment progresser et avancer avec ces baisses de moyens et ces économies de court terme ? Si la France ne veut pas risquer une condamnation européenne pour non-respect de la directive-cadre sur l'eau, il est urgent de réagir.

comment comprendre cette mise en difficulté programmée des agences de l'eau ? L'équation est impossible. Pourtant, l'intérêt des agences de l'eau n'est plus à prouver. Depuis maintenant cinquante ans, ces agences et leurs personnels ont su montrer leur efficacité et leur adaptabilité. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus assumer leurs missions essentielles. Nous sommes tous garants des deniers publics. Bien gérer, c'est prévoir et anticiper. Repousser les problèmes, en limitant les moyens d'étude et d'action, est désastreux pour nos territoires. Pour ces raisons, nous demandons un rapport sur le financement des agences de l'eau. Quel est l'avis de la commission ? J'entends

nous allons lancer une mission interinspections pour clarifier les modalités de financement de la politique de l'eau. Ensuite, nous réunirons des assises de l'eau, auxquelles le Parlement sera naturellement

M. Guillaume Gontard. Nous souhaitons la réalisation d'un rapport sur l'adéquation des moyens et des missions de l'Agence française pour la biodiversité. En effet, au moment de sa création, 225 millions d'euros étaient annoncés pour faire fonctionner cette agence, dont 150 millions provenaient déjà des agences de l'eau. l'eau. Devaient s'y ajouter 60 millions supplémentaires dans le cadre des investissements d'avenir. Au final, dans la loi de finances initiale, ce sont 243 millions d'euros qui ont financé l'AFB. C'était déjà très limité ! Rappelons que les premiers travaux de préfiguration, en 2013, avaient conduit à une estimation des besoins de 400 millions d'euros : nous en sommes loin. L'État, qui versait 34,5 millions d'euros en 2017 pour alimenter le budget de l'agence, ne versera plus rien en 2018. Nous regrettons fortement ce désengagement. La création de l'AFB, agence unique pour la biodiversité, avait pourtant soulevé beaucoup d'espoirs. Au vu des budgets très limités, nous nous demandons aujourd'hui comment l'AFB pourra convenablement remplir ses missions. Nous avons également une opposition de fond sur le principe du financement. En effet, il est regrettable que la seule fiscalité de l'eau, assise sur les redevances des agences de l'eau, finance l'ensemble de la biodiversité, alors que l'AFB exerce sa compétence dans les domaines aquatique, marin et terrestre. Ce financement est également injuste. À travers les agences de l'eau, ce sont les ménages qui seront principalement touchés, puisque 80 % du budget provient des factures d'eau. Le principe, logique et acceptable par tous, selon lequel « l'eau paie l'eau », est détourné, ce qui sera très difficilement accepté et compris par les abonnés.

Il n'y a effectivement pas d'éoliennes en mer, donc le produit de la taxe aujourd'hui est nul. Pour autant, le Gouvernement souhaite avancer vite sur un certain nombre de projets, comme en témoigne l'inauguration, voilà quelques semaines, du projet de parc éolien flottant à Saint-Nazaire. Je ne doute pas que, quand on se rapprochera de la mise en service opérationnelle des éoliennes en mer, il y aura de nouveaux débats sur l'affectation de cette taxe. Dans l'immédiat, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

du 16 février 2017. Il s'agit d'une aide d'un montant de 20 % du prix d'achat, plafonné à 200 euros. Il nous semble important de poursuivre l'effort engagé. Les ventes ont dépassé la barre symbolique des 100 000 unités en 2015, soit Pour 2017, les ventes de VAE s'établiront entre 200 000 et 230 000 unités. Cette hausse de la demande est la preuve que nous sommes non pas en marche, mais en route,

la marche est encore haute, puisque les VAE ne représentent que 3 % des vélos vendus en France. Nous sommes très loin d'autres pays européens comme l'Allemagne. Aussi pensons-nous que ces changements de pratique doivent continuer à être encouragés

En l'occurrence, la commission des finances a choisi de revenir sur le choix initial du Gouvernement, pour les raisons que nous avons évoquées à plusieurs reprises

de proroger ce mécanisme de soutien dans le projet de loi de finances initial, mais, après avoir notamment entendu l'ensemble des acteurs dans le cadre des assises de la mobilité, il lui a semblé important de mettre en place un dispositif nouveau, recentré.

était incompatible avec les aides apportées par les collectivités territoriales. Le dispositif, tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale, répond à ces deux difficultés. D'une part, il place sous conditions de ressources les primes

qui, d'une part, évite les effets d'aubaine en tenant compte des ressources des bénéficiaires, et, d'autre part, vient en appui des politiques menées par les collectivités locales, nous semble approprié et répond aux demandes qui s'expriment dans le cadre des assises de la mobilité. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.

l'avis du Gouvernement ? Le programme spécial 794 a vocation à accompagner des opérations liées à la transition énergétique, notamment l'alimentation de sites isolés l'alimentation de sites isolés à partir des énergies renouvelables. Il a même particulièrement vocation à être mis en oeuvre dans les outre-mer, spécialement pour les communes intérieures en Guyane.